L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à définir les dispositions préalables à une réforme de l'indemnisation des catastrophes naturelles

que nous avons réussi à intégrer l'ensemble des attentes qui avaient été exprimées au Sénat, aussi bien par la commission des finances que par la commission du développement durable. Le texte qui sera adopté cette après-midi permettra notamment de renforcer l'information et l'accompagnement des communes et de leurs administrés, aussi bien avant une catastrophe naturelle que dans la mise en place du dispositif d'indemnisation.

la carte de la sinistralité ou de la potentielle sinistralité du risque retrait-gonflement des argiles révèle que l'ensemble du territoire national pourrait être touché à une échéance de temps

porte de nouveaux équilibres très attendus. J'ai entendu, madame la rapporteure, votre

Qu'il me soit dès lors permis de souligner ici le travail sénatorial sur le thème de la prévention des risques naturels. Face à ces risques et, notamment, à ceux qui sont liés au réchauffement climatique, l'État doit prendre toutes ses responsabilités. Il ne faut pas craindre

Nous nous félicitons également des dispositions visant à permettre la prise en charge des frais de relogement et l'extension de l'indemnisation à l'arrêt des désordres existants, qui sont des mesures utiles et attendues.

de la cellule de soutien. Ensuite, nous comprenons difficilement que la constitution de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles n'ait pas été validée par la commission mixte paritaire, alors même que les partages de connaissances autour des critères de catastrophe naturelle sont souvent jugés aléatoires. Enfin, alors que le Sénat avait permis une prise en compte bien plus importante des phénomènes de retrait-gonflement des argiles à l'article 7,

nous sommes réunis aujourd'hui pour acter une première étape de la réforme nécessaire, voire indispensable, du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Je me réjouis que nous soyons sur le point de franchir cette première étape,

Cette proposition de loi aura mobilisé au total trois commissions permanentes dans les deux chambres du Parlement, autour d'un objectif commun : améliorer la prise en compte des conséquences des catastrophes naturelles dans notre droit.

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, dont j'étais le rapporteur pour avis sur ce texte, avait reçu une délégation au fond pour les articles 2, 4 et 7.

Bien sûr, je suis satisfait de voir que plusieurs évolutions positives vont se concrétiser. Les dispositions de ce texte permettront de renforcer la transparence de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe, de mieux accompagner les communes face à la gestion les communes face à la gestion des événements climatiques exceptionnels et d'améliorer la prise en charge des dommages. J'ai toutefois quelques regrets à la lecture du texte. Mme la rapporteure a pu l'exprimer dans son propos liminaire, j'estime que ce sujet aurait pu et dû être traité plus tôt. Il suffisait à l'Assemblée nationale de se saisir de la proposition de loi de notre collègue Nicole Bonnefoy, quitte à la modifier de façon importante.

Si l'instauration de la prescription quinquennale peut permettre d'améliorer le traitement de certains dossiers, cela me semble quelque peu insuffisant. En outre, j'aurais préféré que certaines dispositions soient maintenues. Je pense notamment à la cellule de soutien pour les maires, dont la création aurait pu être limitée à des événements d'une ampleur toute particulière ou s'inscrire dans une meilleure articulation entre les maires et les préfets, comme nous l'avions proposé. Je pense aussi aux dispositions ajoutées par le Sénat sur le RGA, ou encore à la transparence des travaux de la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, qui aurait pu être plus importante. Je pense enfin aux dispositions relatives à l'information des citoyens à partir d'un point d'entrée unique dématérialisé sur les risques naturels ; il s'agissait pourtant là de concrétiser une annonce de la ministre de la transition écologique ! Je me réjouis cependant que le rôle du référent

je souhaite que nous puissions aujourd'hui valider définitivement ce texte. En effet, malgré des manques et des insuffisances, il comporte des éléments de réponse qui vont vraiment dans le bon sens. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera cette proposition de loi. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous achevons aujourd'hui nos travaux sur le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Je tiens tout d'abord à exprimer ma satisfaction que la commission mixte paritaire, membre suppléant, ait pu trouver un accord sur ce texte aussi important pour les collectivités que nous représentons que pour nos concitoyens sinistrés. Malgré tout, sans surprise, je dresserai un bilan en demi-teinte du parcours législatif de cette proposition de loi d'une part, je regrette que certains apports du Sénat n'aient pas été conservés ; d'autre part, j'estime que le texte aurait pu aller plus loin en matière de protection des sinistrés et d'accompagnement des communes et intercommunalités.

cet accès à un décret n'est pas fait pour nous rassurer, quand on sait le retard pris par la publication de nombreux textes réglementaires d'application des lois. Du point de vue des collectivités, la reprise de la proposition du Sénat de confier au référent départemental, de soutenir les communes déboutées, ainsi que la présence renforcée des élus dans la commission nationale consultative, ou encore l'allongement à vingt-quatre mois du délai pour le dépôt d'une demande de reconnaissance au titre des phénomènes de sécheresse-réhydratation sont des signes positifs et de nature à rassurer nos collègues élus locaux.

Surtout, je regrette le rejet de notre proposition de rendre obligatoire un schéma de prévention des risques naturels majeurs pour les territoires exposés au phénomène du retrait-gonflement des argiles. J'avais souligné en première lecture, lors de la discussion générale, ma sensibilité vis-à-vis de cette problématique, particulièrement saillante dans mon département du Pas-de-Calais. Très clairement, ce texte n'est pas à la hauteur des enjeux ; il n'apportera pas de réelle amélioration face aux situations dramatiques et ubuesques que vivent les sinistrés et les communes concernées. J'éprouve, à titre personnel, une déception forte devant ce rendez-vous manqué, notamment vis-à-vis des familles que j'ai pu croiser.

demande, exprimée notamment par les collectifs de sinistrés, a été exaucée : la communication systématique auprès des assurés des constatations effectuées lors de chaque visite d'experts ; c'est un point essentiel pour des procédures parmi les plus longues. dommage que n'ait pas été maintenu l'apport de notre commission créant un crédit d'impôt pour la prévention des aléas climatiques ; cela aurait pu être une réelle plus-value pour couvrir les dépenses de réduction de la vulnérabilité d'habitations ou de locaux professionnels.

Cela étant, je me félicite que nous progressions globalement sur le sujet sensible de la réparation des dommages consécutifs à une catastrophe naturelle. Mais, parce qu'il y a toujours un « mais », force est de constater que nous sommes encore très en retard quant aux logiques de prévention. Sur ce sujet comme pour d'autres, je pense qu'il nous faut à tout prix engager un travail de fond sur la notion de « coûts évités » et sur l'évaluation de ces derniers. C'est à ce prix que nous pourrons enfin donner à nos actions préventives des moyens dignes de ce nom.

nous sommes aujourd'hui le 16 décembre 2021 : les victimes des aléas climatiques auront donc attendu deux ans pour, enfin, obtenir quelques avancées en matière d'indemnisation des catastrophes naturelles. Je rappelle que, à la suite de la mission d'information sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de nos régimes d'indemnisation, la proposition de loi de notre collègue Nicole Bonnefoy, qui en traduisait les travaux dans un texte législatif, avait été adoptée à l'unanimité par le Sénat en janvier 2020. La suite, nous la connaissons ! Jamais inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ce texte de notre collègue a été repris au travers d'une nouvelle proposition de loi, sur l'initiative d'un député cette fois ; c'est celle dont l'examen touche à son terme

tout par les sinistrés, mais il l'est aussi parce que le temps presse. Le réchauffement climatique n'est plus un concept abstrait, et ses conséquences se font déjà lourdement sentir. Ainsi, depuis 1982, lorsque fut mis en place l'actuel régime des catastrophes naturelles, la quasi-totalité du territoire national a été touchée par un phénomène naturel violent, et bien peu de communes ignorent encore ce qu'est une déclaration de catastrophe naturelle.

Ainsi, le délai de prescription est porté à cinq ans pour les désordres liés à la sécheresse. Les obligations des assureurs sont renforcées, avec par exemple la transmission des comptes rendus de visite à chaque étape de la procédure et l'information apportée aux assurés quant à leurs droits en matière de contre-expertise. De même, la qualité des experts fera maintenant l'objet d'un suivi par la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles, dont le rapport annuel, tout comme celui de la commission interministérielle, sera transmis au Parlement. Enfin, bien que l'idée de la cellule départementale n'ait pas été retenue, le rôle du référent départemental a été clarifié et précisé, pour un meilleur accompagnement des collectivités territoriales et des élus locaux.

Ainsi, la prise en charge des orages de grêles et du phénomène d'échouage des algues sargasses a été retirée du texte. Le crédit d'impôt pour la prévention des aléas climatiques (Cipac) a également été retiré de la proposition de loi. L'instauration de ce dispositif aurait pourtant permis de traiter en amont les conséquences d'un risque climatique croissant. Nous savons tous que le préventif vaut toujours mieux que le seul curatif. Il est ainsi estimé qu'un euro dépensé en prévention permet d'économiser sept euros d'indemnisation. Tout le monde aurait à y gagner : les assurés, les assureurs et les finances publiques. Il est également dommage que ce texte ne traite pas sur le fond le phénomène du retrait-gonflement des sols argileux, lié à la lié à la sécheresse. Nous regrettons vivement la réécriture gouvernementale de l'article 5, qui laisse supposer un affaiblissement de l'indemnisation de cet aléa climatique. Nous prenons cependant acte de la volonté du Gouvernement de créer un régime d'indemnisation à part entière pour les sinistres liés à la sécheresse. En revanche, comme l'a souligné tout à l'heure notre rapporteure Christine il est pour le moins surprenant, voire agaçant, de constater que ce sujet sera traité par le Gouvernement par voie d'ordonnance, à la faveur d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale Jusqu'au bout, le traitement par le Gouvernement des travaux du Sénat, issus de la mission d'information Bonnefoy-Vaspart, aura été bien particulier. Ce texte aurait pu et dû aller plus loin eu égard à l'importance du sujet abordé et aux attentes bien légitimes de nombreux sinistrés.

Au fond, trois mots résument à mes yeux le texte final de cette proposition de loi : transparence, prévention et célérité. Ce texte comporte en effet des avancées juridiques attendues par les sinistrés et beaucoup de collectivités, à commencer par un objectif clairement annoncé depuis le début : mettre fin aux problèmes d'opacité entourant la procédure de reconnaissance des catastrophes naturelles, opacité dénoncée depuis plusieurs années par les élus locaux et les citoyens concernés. Face à ce Face à ce constat, le texte apporte notamment une solution concrète : la nomination d'un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles, référent nommé par arrêté préfectoral dans chaque département. Faciliter les échanges entre les collectivités, les services de l'État et les assureurs, informer davantage les sinistrés, accompagner pour mieux prévenir : telles sont les missions de ce nouveau référent, qui devra répondre aux attentes toujours croissantes en la matière.

sont raccourcis. À compter de la réception de l'accord du sinistré, l'assureur disposera soit d'un délai d'un mois pour des réparations en nature, soit d'un délai de vingt et un jours pour verser une indemnisation pécuniaire D'autre part, le délai pour déposer un dossier de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle passe de dix-huit à vingt-quatre mois, ce qui n'est pas négligeable pour les communes. Ces dernières le réclamaient à juste titre. Le texte comporte d'autres améliorations, notamment sur le risque de sécheresse-réhydratation des sols, un sujet sur lequel nous serons sans doute amenés à échanger à échanger de nouveau. Le dérèglement climatique s'accélère, et ses conséquences sont d'ores et déjà visibles de tous. La sécheresse en est un exemple parmi d'autres. Au cours des vingt dernières années, pas moins de 7 348 désastres naturels ont été enregistrés dans le monde, pour un coût évalué à près de 2 664 milliards d'euros ; c'est presque deux fois plus qu'entre 1980 et 1999 selon un récent rapport du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe. Comme l'a suggéré notre rapporteure, nous avons encore du travail Prévention des risques, élaboration de nouveaux régimes juridiques, protection des sinistrés et de leurs biens : autant de problématiques sur lesquelles nous devrons poursuivre nos réflexions afin d'anticiper l'avenir, l'avenir, de simplifier les procédures et de protéger nos concitoyens. Cependant, des avancées positives sont aujourd'hui face à nous, écrites noir sur blanc. C'est pourquoi le groupe RDPI votera pour l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi. La

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est une règle quasi constante du débat public : le législateur légifère souvent avec un coup de retard. En tant que parlementaires, nous avons tout le loisir de nous en désoler, mais, par construction, il peut difficilement en être autrement : pour agir, nous écoutons d'abord les élus locaux, les spécialistes du domaine, les acteurs qui constatent les problèmes sur le terrain ; toutes ces remontées nous aident, ensuite, à prendre des décisions en adéquation avec le réel. Le dérèglement climatique ne fait pas exception à la règle. Il suffit de discuter avec des assureurs pour savoir qu'il est déjà à l'oeuvre ; leur métier est bouleversé par cette réalité. Voilà plusieurs années qu'ils voient la sinistralité climatique évoluer ; ils ont très bien compris que les règles du jeu ont changé. Nous légiférons, mais le changement opère déjà. Nos agriculteurs et nos viticulteurs l'ont également compris : ils voient leur récolte fluctuer en fonction des aléas climatiques. Pour eux, le dérèglement climatique ressemble à une épée de Damoclès. Les conséquences de ces Les conséquences de ces phénomènes sont lourdes pour le régime assurantiel. En effet, il est désormais bien établi que la fréquence et l'intensité des épisodes climatiques graves sont amenées à augmenter, et avec elles, mécaniquement, les indemnisations versées aux victimes de ces sinistres. Il était donc temps que le législateur se penche à nouveau sur le fonctionnement de ce régime. La multiplication de ces épisodes climatiques, qu'il s'agisse de sécheresses, de gelées ou d'inondations, nous a malheureusement donné de multiples occasions d'identifier les lenteurs et les écueils des procédures liées à la reconnaissance des catastrophes naturelles. Ces lenteurs et ces écueils sont d'autant moins tolérables qu'ils ralentissent et complexifient le versement des indemnisations auxquelles les sinistrés ont droit. Je me réjouis donc que le Sénat et l'Assemblée nationale aient trouvé un accord sur cette proposition de loi visant à définir les dispositions préalables à une réforme de l'indemnisation des catastrophes naturelles. Comme je l'avais déjà dit lors de la première lecture, notre groupe soutient cette démarche, qui va dans le bon sens. Elle rejoint assez largement l'initiative sénatoriale, largement adoptée en janvier 2020, il y a près de deux ans, qui faisait suite à la mission d'information menée par nos collègues Michel Vaspart et Nicole Bonnefoy. Je l'ai dit d'emblée : le législateur agit souvent avec un coup de retard. Cette temporalité l'oblige. Nous n'avons pas de temps à perdre : il était devenu urgent d'améliorer le système. Je me réjouis que les collectivités locales aient pris davantage de place dans la nouvelle mouture du dispositif. Bien sûr, toutes les propositions du Sénat- elles étaient nombreuses sur ce sujet -n'ont pas été retenues ; c'est le jeu de la Commission mixte paritaire. le texte de compromis auquel nos travaux ont abouti améliore substantiellement ce régime assurantiel. C'est une bonne nouvelle, à la fois pour les sinistrés et pour les maires. En effet, les élus locaux et singulièrement les maires se retrouvent le plus souvent en première ligne des opérations. Après la survenue d'un sinistre, en plus des mille services qu'ils rendent à leurs administrés, les maires sont également à l'initiative des procédures qui aboutiront, éventuellement, à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Pourtant, ils se retrouvent souvent démunis face à leurs administrés sinistrés lorsque les décisions tombent et que les motivations manquent. Les maires doivent alors expliquer et justifier une décision qu'ils n'ont pas prise et qu'ils ne comprennent C'est pourquoi il était impératif de rendre la procédure plus lisible et plus transparente pour eux. La création d'un délégué au sein de chaque département pour accompagner les élus dans les démarches à accomplir va dans le bon sens. C'est une réponse concrète pour aider les élus à mieux jouer leur rôle de courroie de transmission entre citoyens sinistrés, d'une part, et administration décisionnaire, d'autre part. Enfin, je regrette que le crédit d'impôt pour la prévention des aléas climatiques, proposé par le Sénat, ne figure pas dans le texte final. Certes, le dispositif n'était peut-être pas suffisamment abouti et il aurait pu représenter un coût très important pour les finances publiques, mais je crois que la piste mérite d'être explorée plus avant. Nous devrons remettre l'ouvrage sur le métier pour élaborer au plus vite un mécanisme opérant. Comme je l'ai dit, nous risquons trop souvent d'agir en retard pour nous permettre de temporiser sur les mesures nécessaires. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants - République et Territoires approuve le texte issu de la commission mixte paritaire, qui apporte de nombreuses avancées et devrait permettre d'améliorer

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Les inondations ont frappé le nord de la France il y a peu. Ces derniers jours, M. le ministre l'a rappelé, ce sont les Pyrénées-Atlantiques et les Landes qui ont été meurtries par des inondations. À l'horizon de 2050, le coût des catastrophes naturelles pourrait croître de 50 % du fait de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements, de l'élévation du niveau de la mer et de la concentration des populations dans les zones à risques. Créé en 1982, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles est un système aujourd'hui dépassé, qui manque de fluidité et de transparence face à une crise climatique qui ne cesse de s'intensifier. C'est un sujet que nous connaissons particulièrement bien au Sénat, et pour cause : le 15 janvier 2020, nous avons adopté à l'unanimité une proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles. Je profite de cette explication de vote pour remercier une fois de plus de leur engagement nos collègues Michel Vaspart et Nicole Bonnefoy, qui ont fourni un travail remarquable et pointé du doigt les difficultés auxquelles est confronté le régime actuel. Il aura donc fallu attendre deux ans de plus pour étudier à nouveau ce sujet, un temps précieux perdu pour les sinistrés et les élus. Je me réjouis néanmoins que nous nous retrouvions aujourd'hui pour voter les conclusions de la commission mixte paritaire et cet accord avec l'Assemblée nationale. Je remercie à ce titre nos collègues Christine Lavarde et Pascal Martin de leur travail important et essentiel, qui a permis au texte final de conserver de nombreux apports du Sénat. Comme vous le savez, les élus sont en première ligne face aux catastrophes naturelles et à leurs conséquences. Ils n'ont eu de cesse de nous alerter sur la nécessité de mieux les informer, les accompagner et les soutenir- cela s'est vérifié dans la vallée de la Roya, comme l'a mentionné Pascal Martin. Je ne Je ne puis que saluer la création d'un référent départemental à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation, qui constitue une réponse concrète à ces demandes et permettra un véritable soutien de proximité pour les communes concernées. D'autres apports du Sénat ont été conservés. Je pense entre autres à la possibilité d'étendre à cinq ans le délai de prescription au cours duquel l'assuré peut exiger de l'assureur le règlement de l'indemnité qui lui est due en cas de sécheresse-réhydratation des sols et de fixer à vingt et un jours le délai dont dispose l'assureur pour verser l'indemnisation due à compter de la réception de l'accord de l'assuré sur le montant. D'une manière générale, cette proposition de loi permet de simplifier les démarches, tout en améliorant la transparence de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et en ouvrant plus de droits aux sinistrés. cette proposition de loi comporte des insuffisances, qui ont d'ores et déjà été évoquées. Je pense au financement du régime des catastrophes naturelles. Ainsi, si le ratio moyen entre sinistralité et primes est de 72 % sur les quinze dernières années, il s'est élevé à 119 % en 2016, 202 % en 2017 et 137 % en 2018, d'après la direction générale du Trésor. Depuis 2016, la sinistralité avoisine 2 milliards d'euros par an,

Cette situation ne peut malheureusement perdurer, et une réflexion sur une nouvelle manière de financer le régime doit être rapidement engagée. Par ailleurs, les mesures relatives au traitement et à l'indemnisation des dommages résultant des mouvements de terrain consécutifs à des phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols argileux ne sont pas à la hauteur des défis. Là encore, des sols argileux ne sont pas à la hauteur des défis. Là encore, le travail doit continuer pour une meilleure prise en compte de ces phénomènes. Bien évidemment, le groupe Les Républicains votera ce texte de compromis qui, malgré ses malgré ses insuffisances, comporte des avancées significatives pour les sinistrés et les élus. Prévention et résilience : le Sénat restera mobilisé pour nourrir les réflexions sur ces sujets. Je suis convaincu que nous aurons l'occasion de nous retrouver dans cet hémicycle pour continuer d'adapter notre pays à ces phénomènes naturels de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. La parole est

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, entre inondations, sécheresses et tempêtes, le nombre des catastrophes naturelles a doublé en vingt ans sous l'effet du changement climatique. Leurs conséquences sont réelles pour beaucoup de nos concitoyens, avec des situations de détresse et de grandes difficultés financières. Ces catastrophes renforcent aussi, il faut le souligner, les responsabilités et sollicitations des élus locaux, qui sont en première ligne pour y faire face. Les difficultés et les défis sont donc nombreux. Nous devons avancer sur les critères de reconnaissance des communes en catastrophe naturelle et sur les rôles respectifs de l'assurance et de l'indemnisation solidaire CatNat, ainsi que préciser mieux les causalités entre les désordres et leurs origines. Des questions très techniques se posent aussi, liées au bâti, à la limite de la garantie décennale de construction, à la comparaison entre les coûts de réparation ou de démolition, au financement des interventions de prévention. La liste est très longue Les conclusions de la commission mixte paritaire sur les dispositions de la proposition de loi ne répondent évidemment pas à toutes ces questions, pas plus qu'à la nécessaire réforme globale de cette indemnisation,

En première lecture, pour éviter que ce texte ne suscite des attentes qui auraient été déçues, j'avais proposé d'en changer l'intitulé, pour signifier que ce texte se situait en amont d'une réforme en profondeur de l'indemnisation des catastrophes naturelles. Le compromis

Je l'ai dit, certaines mesures proposées dans ce texte sont bienvenues, comme la sécurisation de la prise en charge des frais de relogement des personnes sinistrées, ainsi que l'accélération et la simplification des procédures.

face aux événements climatiques provoquant ces dommages importants, même lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la constatation de l'état de catastrophe naturelle. Nous soulignons sur ce point l'accord trouvé sur le périmètre des missions du référent départemental, qui apportera ce soutien aux communes ayant reçu une décision défavorable.

Nous regrettons également la suppression de l'extension du régime de la garantie obligatoire pour cause de tempêtes et catastrophes naturelles pour ce qui concerne les orages de grêle, tout comme la suppression du crédit d'impôt pour la prévention des aléas climatiques. L'article 7 prévoit la remise d'un rapport sur l'opportunité et les moyens d'un renforcement des constructions existantes afin de prévenir les dommages causés par le retrait-gonflement des argiles

Malgré la construction quelque peu baroque de ce texte et d'importantes divergences de fond en matière de responsabilité pénale, la commission mixte paritaire, réunie le 18 novembre dernier à l'Assemblée nationale, a pu aboutir à un accord sur l'ensemble de ces sujets. D'emblée, sur les articles dont s'est particulièrement occupée notre collègue Muriel Jourda, nous avions de nombreux points d'accord. S'agissant des règles relatives à la responsabilité pénale, le Sénat a adopté l'article 2 du projet de loi et considéré que le fait de s'être intoxiqué et d'avoir, dans un état d'abolition du discernement, commis une atteinte aux personnes devait être sanctionné. Cette évolution de notre droit ne va pas de soi, dans la mesure où elle touche à la règle selon laquelle l'état mental de l'auteur d'un acte doit être jugé au moment des faits. nous est toutefois apparu que cette disposition, qui trouve des parallèles dans d'autres pays européens, venait combler une lacune de notre droit. Malheureusement, l'actualité de ces dernières années a montré que c'était nécessaire. adopté l'article 1 , issu des travaux de l'Assemblée nationale, tendant à prévoir que la consommation de drogue ou d'alcool constitue une circonstance aggravante pour les infractions de meurtre, de tortures et actes de barbaries et de violences ayant entraîné la mort ou une mutilation.

Nous avons par ailleurs adopté les dispositions procédurales et celles qui sont relatives aux mineurs délinquants dispositions qui nous ont paru nécessaires et proportionnées. Les mesures tendant à réprimer spécifiquement les violences commises contre les membres des forces à étendre le champ de l'amende forfaitaire délictuelle ou à mieux lutter contre les rodéos urbains ne nous ont pas non plus posé de difficultés. À la suite d'un important travail conduit par nos présidents de commission, nous avons finalement trouvé un accord sur l'article 1 et le champ de l'irresponsabilité pénale. En combinant les rédactions de l'Assemblée et du Sénat, nous aboutissons à un système dans lequel une abolition temporaire du discernement, à la suite d'une intoxication volontaire pour commettre une infraction, entraîne la responsabilité de l'auteur, ce qui nous paraît tout à fait adapté. Dans les cas où l'altération du discernement de l'auteur de l'acte résulte de son propre fait, le juge du fond se prononcera à huis clos, ce qui correspond à la volonté du Sénat de ne pas créer de « justice spectacle Il me semble que cette position d'équilibre répond à la volonté d'avoir un procès qui détermine clairement les responsabilités, sans toucher aux fondements de notre droit pénal.

Les articles relatifs au contrôle des armes à l'échelon national contiennent des évolutions de bon sens, permettant une meilleure effectivité des interdictions d'acquisition et de détention et un plus grand contrôle de l'accès aux métiers de l'armurerie et de l'armement. Nous leur avons apporté quelques précisions, que les rapporteurs pour l'Assemblée nationale ont acceptées. Plusieurs articles reprenaient ensuite des dispositions de la loi Sécurité globale ayant fait l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel. Il s'agissait tout d'abord de l'article 6, qui vise à accompagner la montée en puissance de la réserve civile de la police nationale. Reprise d'un amendement sénatorial inséré dans dans la proposition de loi relative à la sécurité globale, l'article ne soulevait pas de difficulté entre nos deux assemblées. J'en viens à la captation d'images par les forces de sécurité. Plusieurs articles du projet de loi proposent de donner aux policiers et aux gendarmes les moyens de mieux tirer parti des nouvelles technologies de captation d'images. Le Sénat s'est attaché à trouver un équilibre entre opérationnalité de l'usage des caméras et protection du droit au respect de la vie privée. Nous avons également choisi d'ouvrir l'usage des drones aux polices municipales, comme nous l'avions fait au mois de mars dernier, et de donner à l'usage des drones en matière judiciaire un cadre législatif, suivant en cela l'avis rendu au cours du mois d'octobre dernier par le Conseil d'État. Deux points que nous avons ajoutés posaient plus particulièrement problème aux rapporteurs pour l'Assemblée nationale. Il s'agissait notamment de la durée de conservation des enregistrements issus de la surveillance des cellules de garde à vue, que nous avions allongée pour permettre l'exercice des droits de la défense, et des modalités de consultation des images captées par des caméras aéroportées.

administratives et disciplinaires, d'une meilleure information des personnes dont l'image est captée ou de la consultation des images issues des caméras embarquées par les agents eux-mêmes. Mes chers collègues, il me semble donc que l'accord que nous vous proposons d'adopter aujourd'hui constitue une position d'équilibre entre nos deux assemblées. Nous nous en réjouissons.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureuse de vous retrouver à la suite de l'accord trouvé sur ce texte important par la commission mixte paritaire réunie le mois dernier et de représenter le Gouvernement devant la Haute-Assemblée. Comme l'a rappelé Éric Dupond-Moretti, le 14 avril dernier, la Cour de cassation confirmait la déclaration d'irresponsabilité pénale du meurtrier de Mme Halimi, reconnaissant que l'auteur avait agi sous le coup de l'abolition de son discernement, tout en consacrant le caractère antisémite de ce meurtre. Cette décision a provoqué un profond et très légitime émoi et un sentiment d'incompréhension. Elle a pourtant respecté l'état actuel de notre droit : même lorsqu'une personne mise en cause a provoqué elle-même la perte de son discernement, elle ne peut répondre devant la justice des actes qu'elle a alors commis. Cette impossibilité de distinguer l'origine de la perte de discernement n'est plus acceptable. Tel a été le sens des propos du Président de la République au mois d'avril dernier. mixte paritaire, la loi permettra, comme nous nous y étions engagés, la distinction entre un individu atteint d'une pathologie psychiatrique qui le prive de tout libre arbitre et celui qui doit sa folie à la consommation volontaire de produits psychotropes. Il était impératif de ne pas de ne pas laisser ces situations perdurer, mais aussi, je me dois de le rappeler, de respecter toutes les précautions, notamment constitutionnelles, que requiert la délicate évolution du régime de la responsabilité pénale. Le texte issu de la commission mixte modifier le régime de l'irresponsabilité pénale dans le respect le plus absolu de nos exigences constitutionnelles. Le nouvel article 122-1-1 du code pénal prévoit ainsi que celui qui s'est volontairement intoxiqué dans le but de commettre une infraction ne pourra plus bénéficier du régime de l'irresponsabilité pénale si l'abolition de son discernement résulte directement de cette consommation. La loi a également été modifiée, afin que la déclaration d'irresponsabilité pénale, dans le cas exclusif d'avis divergents des expertises psychiatriques, relève désormais de l'appréciation des juges du fond, et non plus uniquement de celle du magistrat instructeur. C'est le tribunal correctionnel ou la cour d'assises qui statuera, lors d'une audience à part et se déroulant à huis clos, sur la question de la responsabilité pénale du mis en cause et de sa capacité à répondre de ses actes devant les juges. L'ensemble de ces dispositions respectent la ligne rouge que nous avions tracée : on ne juge pas et on ne jugera jamais les fous. Cette loi permettra de poursuivre et de juger des actes qui n'étaient auparavant pas sanctionnables. En effet, avec la création d'infractions autonomes spécifiques, ce texte vient combler une lacune juridique majeure, comme l'avait indiqué l'avocate générale de la Cour de cassation dans ses conclusions. Ces nouveaux délits puniront, pas l'acte commis en état d'abolition temporaire du discernement, mais bien la consommation fautive et volontaire de psychotropes qui l'a précédé. La commission mixte paritaire a dressé la liste limitative des infractions susceptibles de donner lieu à des poursuites sur ce fondement, retenant les homicides volontaires, les viols, les actes de toitures et de barbarie,

commis à l'encontre de toutes les professions qui, dans l'espace public, assurent notre sécurité au quotidien. La protection des policiers, gendarmes, militaires de l'opération Sentinelle, douaniers, agents pénitentiaires, policiers municipaux, gardes champêtres et pompiers sera renforcée, car il n'est plus tolérable que leur que leur engagement au service de la collectivité les érige en cible. Le message est simple : nous protégeons ceux qui nous protègent. Ce projet de loi comporte par ailleurs des avancées procédurales souhaitées par les acteurs judiciaires, lorsqu'ils sont confrontés à des délinquants refusant toute identification. L'effectivité de la loi pénale nécessite d'établir efficacement une identité judiciaire. Nous avions la responsabilité de renforcer le cadre procédural de cette identification. Désormais, les enquêteurs pourront recourir à la prise d'empreinte sous contrainte dans le cadre d'un dispositif équilibré intégrant des garanties renforcées à l'égard des mineurs. Désormais, la juridiction improprement saisie sur le fondement de l'âge de l'auteur pourra placer en détention le majeur ou le mineur, afin de le présenter devant la juridiction compétente dans des délais très courts. La procédure pénale actuelle permettait de remettre en liberté des prévenus à la suite de la déclaration d'incompétence de la juridiction ; cela ne sera plus le cas. Il s'agit là de garantir l'effectivité de la loi pénale. Nous le devons bien sûr aux victimes, nous le devons aussi aux vrais mineurs, qui pourront ainsi bénéficier des dispositifs éducatifs adaptés à leur âge.

Lorsqu'elles sont sur nos routes, nos forces de sécurité subissent de plus en plus le danger représenté par le refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. À ce titre, le projet de loi renforce les mesures conservatoires et le régime des peines applicables.

L'article 18 du projet de loi vise ainsi à faciliter l'identification des auteurs de ces infractions et à empêcher la restitution de véhicules. En matière d'infractions routières, l'article 17 étend la liste des infractions au code de la route qui peuvent être constatées par les gardes particuliers.

Cela passe par la création d'une réserve opérationnelle, qui permettra à la police nationale de disposer de plus de réservistes issus de la société civile pour renforcer l'action des policiers. Ce projet de loi permet également de compléter les moyens à disposition de nos forces de l'ordre. La captation d'images est aujourd'hui au coeur de l'action des forces de sécurité, compte tenu de son utilité opérationnelle. Toute l'attention doit être portée à l'équilibre entre l'intérêt opérationnel des forces de sécurité et la préservation des droits et libertés fondamentaux. Le Gouvernement a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi pour une sécurité globale et préservant les libertés ; il en tire les conséquences dans ce projet de loi. Ce texte permet ainsi la définition d'un cadre juridique solide, autorisant la captation d'images depuis des dispositifs vidéo installés sur des aéronefs, avec ou sans personne à bord. Il offre ainsi les garanties nécessaires, tout en permettant à nos forces de sécurité de disposer d'outils efficaces. Le Sénat a également introduit dans ce projet de loi une expérimentation permettant aux polices municipales d'utiliser des drones, si l'ensemble des garanties nécessaires sont réunies et sous réserve que ces polices visent un champ clairement défini de finalités proportionnées à l'égard de l'usage d'une telle technologie. concerne l'usage des captations d'images par des engins aéroportés à des fins judiciaires, le Conseil d'État confirmé, dans un avis rendu le 12 octobre dernier, la nécessité de légiférer. commission mixte paritaire prévoit que l'usage judiciaire de ces dispositifs de captation d'images dans l'espace public puisse être autorisé en cas de crime ou délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, en cas de procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition, ou encore en cas de recherche d'une personne en fuite. Ces captations devront être préalablement autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Le texte comporte également un dispositif pour les caméras embarquées dans les véhicules des services de l'État.

de garde à vue, avec pour objectif de diminuer les risques de suicide, d'automutilation, d'agression ou d'évasion. Toutefois, la captation d'images dans les cellules de garde à vue ne saurait être systématique et de durée indéterminée. ce point, le texte issu de la CMP est équilibré, du point de vue tant des garanties applicables au dispositif que des durées de conservation des enregistrements vidéo au regard de leur finalité.

paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par

Mais, finalement, le dispositif adopté ne fait qu'entériner la jurisprudence. L'aggravation des peines pour utilisation de stupéfiants et

dont le consentement a été aboli. Le rapport Houillon estime que les mesures de sûreté sont trop limitées et notamment ne permettent pas à la juridiction d'ordonner des soins psychiatriques sans consentement, sauf hospitalisation complète. Il y a là une faille dans le dispositif, et nous devrons travailler à une judiciarisation des mesures d'hospitalisation et de contrôle. J'avais interrogé le garde des sceaux

par une mesure d'irresponsabilité à un moment ou à un autre. Or ces 15 000 personnes ne sont pas suivies. Elles sont dans la nature, sans aucun

dans des dispositifs parfois exigeants et souvent complexes, les conditions garantissant à chacun sa sûreté, sa sécurité, sa sérénité et,, l'exercice paisible de sa liberté. En premier lieu, il y a la question de l'irresponsabilité pénale, tristement mise en exergue par le meurtre de Sarah Halimi. Il faut redire que notre assemblée s'était montrée sensible très tôt aux difficultés pouvant exister dans le lien entre psychiatrie et droit pénal. Dès avant la décision de la cour d'appel de Paris dans l'affaire Halimi, le Sénat avait ainsi constitué, dès le mois de juillet 2019, un groupe de travail commun entre sa commission des affaires sociales

Nous avons travaillé, notamment nos rapporteurs, afin que cela ne se reproduise pas. J'espère donc que ce nouveau texte ne butera pas une nouvelle fois sur les juridictions.

Toutefois, nous regrettons leur disparition du texte, car ils y traitaient de points particulièrement importants. Je pense notamment aux articles 3 B, 4 3 B, 4 et 7 . L'article 3 B, traitant des mesures pouvant être ordonnées par le juge après que l'irresponsabilité pénale ait été constatée, répondait à une attente consensuelle des praticiens. Il autorisait la juridiction à ordonner des soins psychiatriques sans hospitalisation complète. La souplesse de ce dispositif permettait au droit de mieux s'adapter à la pratique des juges et des médecins. L'argument qui nous fut présenté par le Gouvernement lors de notre examen en séance publique fut de dire que le juge n'est pas médecin Dont acte, mais il demeure que le code de procédure pénale lui permet d'ordonner l'admission en soins psychiatriques de la personne irresponsable, sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est difficile d'y voir autre chose qu'une décision médicale ... Dès lors, pourquoi ne pas lui laisser la possibilité d'en prendre d'autres ? Je me permets également de revenir sur l'article 4 , que notre hémicycle avait adopté et qui concernait l'anonymisation des témoins d'agressions de sapeurs-pompiers. Chacun entendra l'argument selon lequel ce dispositif serait déjà satisfait, dans la mesure où il n'y aurait que peu de cas de violences exercées contre des pompiers qui soient punis de moins de trois ans d'emprisonnement. Il demeure que le sujet est gravissime et que, dès lors, il ne faut pas craindre d'inscrire dans la loi, même symboliquement,

Sainte-Barbe ... Le groupe RDSE regrette donc la disparition de ce dispositif. Enfin, l'article 7 , adopté par notre assemblée, prévoyait la remise au Parlement par le Gouvernement d'un rapport détaillant les grands axes de la politique globale de réhabilitation des cellules de gardes à vue. Cette demande de rapport avait été adoptée malgré la jurisprudence constante de notre assemblée, qui n'aime pas les rapports. Je crois qu'elle aurait pu être maintenue afin de dresser un état des lieux sur cette question. C'est un sujet pour lequel il faut de la transparence, à la fois pour améliorer les conditions d'accueil des individus gardés à vue et pour dire, le cas échéant, quand les cellules ne sont pas dans un état indigne. Bien entendu, ces regrets ne nous empêcheront pas de voter ce projet de loi.

était parti à Poitiers. Il devait aller entendre un discours de M. le Président de la République, qui ouvrait, en fin de mandat, les États généraux de la justice.

Je ne tiens pas à faire preuve ici d'un quelconque triomphalisme politicien. Le budget de la justice n'a pas suffisamment augmenté depuis très longtemps. Il est vrai qu'il a progressé de 8 % cette année, comme l'année précédente, mais nous voyons bien que nous sommes loin du compte.

-il est nécessaire de prendre en compte la situation dans laquelle une personne choisit elle-même d'organiser son absence de discernement.

S'il n'y avait eu que cette partie du texte, nous aurions voté pour, en dépit des quelques remarques que je viens de faire. Dommage ! En revanche, pour ce qui est de la seconde partie, portant sur la sécurité, nous sommes bien sûr

d'un autre texte. Cela dit, certaines mesures sont revenues parce que le Conseil constitutionnel les avait critiquées. Nous persistons à dire que nous sommes en désaccord avec les mesures relatives aux drones et à la vidéosurveillance

Les Français ont été nombreux à ne pas comprendre la décision rendue par la justice dans l'affaire Sarah Halimi. Cette incompréhension ne doit cependant pas laisser croire que les juges ont failli. Il faut le dire ici, ils ont parfaitement appliqué la règle qui était inscrite dans notre droit. C'est bien la règle fixée qui était en cause et que beaucoup ont souhaité voir modifier.

Désormais, ceux qui s'intoxiquent en vue de commettre un crime ou un délit devront répondre de cette intoxication, dès lors qu'elle aura été suivie d'une infraction. Une consommation volontaire de substances psychoactives, entraînant l'abolition du discernement, ne sera plus synonyme d'irresponsabilité pénale. Nous soutenons ces dispositions, tout comme nous soutenons le message qu'elles envoient l'intoxication volontaire n'est pas exonératoire de la responsabilité pénale. Nos concitoyens doivent savoir que ces consommations sont des actes répréhensibles en tant que tels, qui seront punis à ce titre. Dans cette perspective, nous nous félicitons que ce texte inscrive dans notre droit la consommation volontaire d'alcool ou de stupéfiants comme une circonstance aggravante de l'infraction. Cette disposition est la contrepartie nécessaire de la responsabilité civile des individus : chacun doit répondre de ses actes, ainsi que de ses consommations. Les articles concernant la responsabilité pénale sont les plus emblématiques de ce texte, mais celui-ci comporte bien d'autres avancées, portant sur la sécurité au quotidien de nos compatriotes. Les confiscations et les destructions de véhicules ayant été utilisés pour commettre des rodéos urbains, dont on entend régulièrement seront désormais facilitées. C'est une réponse de fermeté que nous soutenons et qui est attendue par les riverains. Nous nous félicitons également de l'extension de la procédure d'amende forfaitaire aux vols de faible valeur. Cette procédure, qui a fait ses preuves, préserve les droits des victimes en imposant la restitution de l'objet ou l'indemnisation de la victime. Ne pensons pas que la faible valeur de ces vols les rende anecdotiques : ils font partie de ces infractions du quotidien qui empoisonnent la vie de nos concitoyens. L'amende forfaitaire permettra d'apporter une réponse rapide et proportionnée à ces délits. Le texte comporte également toute une série de dispositions visant à renforcer la protection de nos forces de l'ordre. Il est nécessaire de protéger ceux qui nous protègent, parfois au péril de leur vie. Nous soutenons donc le renforcement des sanctions portant sur les violences commises contre les policiers, les gendarmes et les membres de leur famille. Ceux qui s'attaquent à eux doivent savoir qu'ils s'attaquent à la République et qu'ils seront punis en conséquence. Il fallait enfin permettre aux forces de l'ordre d'utiliser les moyens vidéo modernes, pour mener leurs enquêtes, mais aussi pour protéger les gendarmes et les policiers engagés dans des opérations de terrain. Ces dispositions permettront d'embarquer des caméras sur les véhicules, mais aussi sur des drones. Mon collègue du Nord, Jean-Pierre Decool, s'associe à moi pour saluer tout particulièrement l'article 8, qui ouvre l'utilisation de drones à la lutte contre l'immigration irrégulière,

Mais leur utilisation ne pouvait pas se faire au détriment des libertés individuelles. Le texte reprend par conséquent plusieurs recommandations formulées par la CNIL à cet égard.

L'accord obtenu sur le premier volet, le plus débattu de ce texte, a permis de répondre à la vive émotion suscitée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation, au mois d'avril dernier, prononçant l'irresponsabilité pénale de l'auteur du meurtre de Sarah Halimi. Ce sujet d'actualité renvoie à un débat qui agite la communauté juridique en particulier, et l'opinion publique en général, depuis fort longtemps : doit-on, ou non, juger les fous ? Le 18 novembre dernier, nos deux chambres se sont accordées sur la possibilité- inédite -de poursuivre et de condamner celui qui se serait intoxiqué et aurait commis une atteinte grave aux personnes dans un état d'abolition temporaire du discernement. Les membres de la commission mixte paritaire ont néanmoins pris soin d'apporter plusieurs garanties indispensables à cette nouvelle procédure, que notre groupe salue, en particulier l'exigence préalable d'expertises psychiatriques contradictoires. Nous nous félicitons également de ce que le Sénat ait obtenu gain de cause sur un point qui nous tenait particulièrement à coeur, celui de la compétence de la juridiction de jugement pour la déclaration d'irresponsabilité. qui était prévu dans le texte initial, la déclaration d'irresponsabilité sera prise par le tribunal correctionnel ou par la cour d'assises, au terme d'un procès. Alors que le texte initial confiait cette compétence à la chambre de l'instruction, cette modification substantielle octroie aux victimes un cadre symbolique s'il en est leur permettant, en outre, de mieux comprendre les raisons pour lesquelles une personne mise en cause peut être déclarée irresponsable par les juges du fond. Cette disposition nous semble de nature à éviter les incompréhensions pleinement légitimes des victimes, et parfois leur indignation, à laquelle nous nous associons. Le volet sécuritaire de ce projet de loi comporte des avancées bien réelles. Il en est ainsi du renforcement du contrôle des armes au plan national, de l'accompagnement de la montée en puissance de la réserve civile de la police nationale ou encore du meilleur encadrement de la captation d'images par les forces de sécurité. Nous tenons toutefois à exprimer un regret, relatif à l'abandon des dispositions de la proposition de loi du président Kanner, qu'a souligné également le président Requier. C'est vrai ! Ces dispositions visaient à étendre le dispositif qui anonymise l'identité des témoins aux procédures portant sur les infractions commises sur un sapeur-pompier. Elles avaient pourtant été adoptées à l'unanimité au Sénat, il y a déjà deux ans. Malgré cela, nous nous félicitions de l'accord obtenu, et je ne doute pas qu'une grande majorité de notre groupe se prononcera en faveur de ce texte, dans la rédaction issue des travaux de la

Sa première partie est guidée par la volonté de modifier les conditions de la déclaration d'irresponsabilité pénale. Ce principe à valeur constitutionnelle est pourtant, comme le rappelle le Conseil d'État dans son avis, « l'un des fondements anciens et constants du droit pénal », car « il ne peut y avoir de responsabilité sans libre arbitre Ce projet de loi s'inscrit dans la lignée des travaux de notre assemblée, qui entendaient déjà répondre à ce qui avait été compris par beaucoup comme un appel du pied de la Cour de cassation. La loi ne distingue pas selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition du discernement. Mais la CMP a abouti à un texte qui permet en réalité d'écarter l'application de l'ensemble de l'article 122-1 du code pénal si l'abolition du discernement résulte d'un fait fautif antérieur, à savoir si, « dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction commettre l'infraction ». Je le redis : sauf à promouvoir une théorie de la folie volontaire, cette vision est trop réductrice et ne trouve pas écho auprès des professionnels du droit et de la médecine ! Certes, un comportement volontaire peut directement contribuer au déclenchement de l'abolition du discernement,

pourquoi avoir limité le fait fautif à la prise de substances psychoactives ? Même à considérer qu'il faille distinguer entre abolition volontaire ou non et que chacun ait une connaissance assez fine de son état de santé et des effets de chacune de ses consommations, pourquoi limiter l'exception à la prise volontaire de substances psychoactives ? Pourquoi, par exemple, ne pas prendre en compte également l'arrêt de la prise de certaines substances ? Cela n'a pas de sens

Notre groupe regrette aussi profondément que le Gouvernement refuse encore une fois de donner les moyens aux experts psychiatres de poursuivre leur mission de diagnostic et d'expertise dans des conditions plus adaptées à leurs missions. Que dire maintenant de la deuxième partie du texte, aussi sécuritaire qu'électoraliste ? Le projet que vous nous présentez comporte notamment de nouveaux délits autonomes visant à réprimer les violences commises sur nos forces de sécurité. Si nous condamnons encore et toujours ces violences, la qualité de « dépositaire de l'autorité publique » est déjà une circonstance aggravante qui permet l'application de peines plus lourdes. Pour des gens qui fustigent souvent les postures victimaires ou la concurrence des douleurs, je vous trouve bien réceptifs aux revendications de certains syndicats

La Défenseure des droits appelle à une plus grande vigilance face à un texte dont le manque de précision compromet l'effectivité de la restriction de l'application de la vidéosurveillance, et qui pourrait conduire à la systématisation L'article 8 porte sur l'utilisation de caméras embarquées sur des drones ou tout autre aéronef. Là encore, des mesures censurées par le Conseil constitutionnel nous reviennent dans une version prétendument mieux cadrée.

Notre groupe s'oppose à ces dispositions liberticides. De manière générale, nous prendrons nos responsabilités face à ce que nous considérons comme une attaque caractérisée contre l'équilibre de notre société. Nous jouerons notre rôle de gardien des valeurs républicaines et constitutionnelles. C'est pourquoi

Premièrement, ces conclusions actent une exception d'irresponsabilité pénale. Pour l'Assemblée nationale, c'est le cas lorsque l'abolition temporaire du discernement résulte de la consommation proche ou volontaire de psychotropes dans le but de commettre une infraction.

conséquences non négligeables et fait notamment émerger la notion d'« abolition temporaire liée à un fait fautif ». Je vous le redis, légiférer en ce sens, ce serait oublier que ces comportements ne sont pas nécessairement fautifs et qu'ils peuvent être, non pas la cause

pour notre part, comme l'a souligné le rapport Houillon-Raimbourg, que « l'abolition du discernement au moment de l'acte est exclusive de l'intention au sens du droit pénal [ ...] et qu'il ne peut être transigé avec ce principe sans remettre en cause notre édifice pénal

particulier l'autorisation des captations vidéo dans les locaux de garde à vue ou des drones et caméras embarqués dans les véhicules de police. Le texte final ouvre également l'usage des drones aux policiers municipaux,

ces mesures de sécurité intérieure- à l'exception de quelques-unes, comme le contrôle de la détention d'armes, qui sont positives -nous renvoient à un modèle de société dont nous ne voulons pas : une société de la surveillance de tous, partout, tout le temps, dans la droite ligne de la logique répressive et sécuritaire développée ces dernières années. Je déplore l'adoption conforme par notre assemblée de l'article 16 de ce projet de loi, qui stigmatise encore un peu plus les mineurs non accompagnés, en permettant de procéder, malgré leur refus, à un relevé de leurs empreintes digitales ou palmaires ou à une prise de photographie lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis un crime ou un délit. Cet article s'inscrit dans le climat

Il marque l'aboutissement de travaux approfondis, à l'occasion de l'examen de plusieurs textes successifs. Le régime d'irresponsabilité pénale des personnes dont le discernement est aboli lors de la commission d'une infraction du fait de la consommation délibérée de substances psychoactives psychoactives avait ainsi fait l'objet au Sénat, sur l'initiative notamment de notre collègue Nathalie Goulet, d'un débat et d'une proposition de loi. D'autres dispositions du texte, relatives notamment aux régimes de captation d'images, tirent les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, qui avait précédemment fait l'objet d'un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Cet aboutissement marque également celui des engagements de l'exécutif, après les décisions de justice successives rendues dans l'affaire du meurtre de Sarah Halimi, jusqu'à la décision de la Cour de cassation en avril dernier, et les violences commises à l'encontre des forces de sécurité. Cet aboutissement marque enfin une convergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat, après une commission mixte paritaire dont le groupe RDPI salue pleinement l'issue favorable et les évolutions importantes qu'elle permet.

L'affaire Halimi et la sidération légitime qu'elle a suscitée l'ont rappelé avec gravité. Le projet de loi marque sur ce point une évolution majeure de notre droit pénal, dans le respect des exigences constitutionnelles et sans remettre en cause le principe selon lequel « on ne juge pas les fous L'article 2 avait dès la première lecture fait l'objet de l'approbation de nos rapporteurs. Il comble une lacune de notre droit en permettant de poursuivre et de juger spécifiquement la consommation volontaire de substances psychoactives ayant entraîné une abolition temporaire du discernement sous l'empire de laquelle ont été commises certaines atteintes à la vie ou à l'intégrité de la personne, de même de même qu'un viol. La CMP a ensuite permis de trouver un équilibre au sein de l'article 1. Celui-ci permettra donc, comme le souhaitait le Gouvernement, avec le soutien de notre groupe notamment, d'écarter l'irresponsabilité pénale d'une personne qui s'est volontairement intoxiquée afin de commettre un crime ou un délit. Cet article modifie également les modalités de déclaration d'irresponsabilité pénale d'une personne dont l'abolition du discernement résulte de son fait, comme l'avait souhaité notre rapporteur. est ainsi mieux encadré, dans le respect des exigences de notre État de droit : le renvoi de cette question aux juges du fond est limité à l'existence d'expertises psychiatriques divergentes et soumis à huis clos. Notre groupe salue par ailleurs l'accord trouvé sur les dispositions relatives à la sécurité intérieure, notamment sur les différents régimes de vidéoprotection, qui faisaient l'objet d'une convergence de fond dès la première lecture. Je m'arrêterai un instant sur les drones. Le Conseil constitutionnel avait rappelé qu'il nous était loisible d'autoriser la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par drones aux fins notamment du maintien de l'ordre et de la sécurité publics. Le texte soumis aujourd'hui à notre ultime approbation contient les garanties supplémentaires qui étaient nécessaires pour assurer une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l'ordre public et le droit au respect de la vie privée. Nous saluons également la reprise dans ce texte de l'extension aux polices municipales de la faculté d'utiliser des drones, portée par notre collègue Alain Richard avec le soutien du Gouvernement au sein d'un précédent texte de loi. J'aurais pu m'arrêter, aussi, sur le renforcement de la répression des violences commises à l'encontre des forces de sécurité intérieure, de l'encadrement de la détention d'armes, ou de la lutte contre les rodéos motorisés et les refus d'obtempérer. Autant de dispositions utiles pour agir contre la criminalité et protéger tous nos concitoyens, dans une approche exigeante et équilibrée en matière de droits et libertés. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera ce texte. Conformément